L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

Ainsi, votre proposition de déterminer par décret les missions des délégations départementales des ARS me semble trop rigide ; en outre, cela ne En effet, encadrer dans un texte de niveau réglementaire les missions de ces délégations départementales n'est pas souhaitable, tant leurs situations et les besoins des territoires sont divers. Il est nécessaire de conserver une forte capacité d'adaptation et de réactivité. Le Gouvernement propose plutôt un document souple, comme une charte, qu'il n'est pas nécessaire de prévoir dans la loi.

le projet régional de santé fait d'ores et déjà l'objet d'importantes consultations avant d'être arrêté par le directeur Il est publié après avis du conseil de surveillance et après consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie, du préfet de région et des collectivités territoriales de la région.

au-delà de sa fonction de direction de l'ARS, il est aussi investi de prérogatives qu'il exerce en tant que dépositaire d'un pouvoir d'État. Les fonctions de police sanitaire, qui intègrent la responsabilité d'arrêter le projet régional de santé, participent de cette catégorie et ne peuvent donc relever du conseil d'administration

un désaccord entre deux présidents étant susceptible de bloquer le fonctionnement de l'agence. Par ailleurs, le conseil régional ne dispose pas, en matière sanitaire, de compétences qui justifieraient cette coprésidence. une présidence par le préfet de région est justifiée par la nécessité de garantir la cohérence de l'action de l'ensemble des services et des opérateurs de l'État. Tel est bien le souhait que j'avais entendu, tant présent amendement tend enfin à supprimer la disposition prévoyant que les représentants de l'État ne peuvent disposer de plus de voix que les représentants des collectivités au sein du conseil d'administration. la composition détaillée du conseil d'administration relève du niveau réglementaire. Le Gouvernement sera toutefois attentif à la répartition des sièges entre trois groupes d'acteurs : les administrations, c'est-à-dire l'État et l'assurance maladie,

du conseil de surveillance de l'ARS en conseil d'administration, ni sur le renforcement de la place des élus, qui est à notre sens fondamental. Merci

ARS. Actuellement, ces élus ne disposent que de quatre ou cinq voix face aux douze voix des représentants de l'État et aux neuf voix de l'assurance maladie. Il apparaît d'autant plus pertinent de renforcer considérablement le poids des élus dans les conseils d'administration des ARS

le délégué départemental de l'ARS relève de l'autorité fonctionnelle du directeur général de l'agence, lui-même nommé en conseil des ministres.

la compétence régalienne de l'État en matière de santé. Toutefois, on a bien constaté que l'ARS seule n'est pas en capacité d'agir si le bras armé que représentent les collectivités n'est pas mobilisé.

le Gouvernement propose d'élargir la compétence des collectivités en matière de santé, en leur donnant la possibilité de financer des établissements.

l'échelon départemental des ARS doit prendre de l'importance et refuser d'en définir le cadre. Nous sommes dans une République de l'écrit, malgré tout. Il est donc temps de mettre autour de la table les associations d'élus, les professionnels de santé et tous ceux qui sont concernés par ce sujet

des délégués départementaux des ARS n'ont pas été recrutés au bon niveau et n'ont pas toujours

Il est donc proposé au travers de cet amendement que, au sein du conseil d'administration de l'ARS, puisse siéger un élu représentant les secteurs de montagne, désigné par le comité de massif. Les comités de massif ont, depuis longtemps, fait la preuve de leur efficacité en matière de gestion, notamment de service en montagne, ce dernier portant une spécificité particulière. Leur parole doit pouvoir être portée au sein des conseils d'administration des ARS.

à garantir la présence d'un représentant d'une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d'administration des ARS. La

Cet amendement vise à garantir la présence d'un représentant d'une collectivité ou groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d'administration des agences régionales de santé, afin de s'assurer de la prise en compte des spécificités des territoires de montagne.

Dans les régions concernées, la représentation des zones de montagne pourrait être intéressante, mais il n'y a pas de sens à la généraliser. Laissons à chaque région la possibilité de s'organiser en fonction

Dans le cadre de la régulation de l'offre de soins, les agences régionales de santé pilotent les politiques de santé publique dans nos territoires. Cet amendement tend à proposer que les présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, siègent au sein des conseils d'administration des ARS, afin qu'ils puissent prendre part aux décisions qui les affecteront de manière directe. Il existe des interactions constantes entre les services d'incendie et de secours et les ARS. Ces dernières portent notamment sur la participation des services d'incendie et de secours à l'aide médicale urgente, mais aussi en matière de coopération des transports sanitaires.

des affaires sociales ? La composition actuelle du conseil d'administration des ARS ouvre déjà la possibilité de représenter les services d'incendie et de secours participant aux secours et soins d'urgence, ou, à tout le moins, de porter leur voix.

Genet, pour présenter l'amendement n° 201 rectifié Le présent texte étend les missions du conseil d'administration des ARS, qui fixe les grandes orientations de la politique menée par l'agence, en ce qui concerne la conclusion et l'exécution de conventions avec les collectivités territoriales pour la mise en oeuvre du projet régional de santé. L'objet de cet amendement est de compléter les missions du conseil d'administration des ARS : celui-ci doit statuer sur toutes les décisions prises en matière d'offres de soins. n° 1013 rectifié. Afin qu'aucune décision en matière d'offres de soins n'échappe au conseil administration des ARS, il est proposé ici d'étendre le champ d'action de ce dernier, pour qu'il statue sur toutes les décisions concernant l'offre de soins.

La question de la désertification médicale des territoires est au coeur des enjeux sanitaires de notre pays. De nombreuses réflexions ont été menées à ce sujet, sans pour autant déboucher sur des solutions pérennes. Aussi, il est nécessaire que tous les acteurs du milieu de la santé soient mobilisés, afin de lutter efficacement contre ces déserts médicaux. Naturellement, cela doit également concerner les agences régionales de santé et, plus particulièrement, leurs organes de gouvernance. projet de loi propose que les conseils de gouvernance des ARS deviennent des conseils d'administration. Cet amendement vise donc à inscrire, parmi les missions de ce nouveau conseil, celle de dresser un bilan de l'état territorial de la désertification médicale, ainsi que de proposer d'éventuelles solutions pour y remédier. Jean-Yves Roux et les auteurs de cet amendement insistent sur le fait que les régions, parfois très grandes, ne permettent pas de prendre des solutions adaptées aux différentes situations observées, mais aussi aux initiatives ou aux orientations locales en matière d'organisation de santé publique.

discuté ici. Toutefois, il n'appartient pas à un conseil d'administration d'effectuer un état des lieux de la désertification médicale, qui est réalisé, par ailleurs, par l'ARS, dans le cadre des zonages. par ailleurs, par l'ARS, dans le cadre des zonages. Au niveau du conseil d'administration, les réponses à apporter aux enjeux d'accès aux soins sont déjà couvertes par les discussions dans le cadre du projet régional de santé et pourront être abordées dans le bilan d'exécution, en particulier des crédits des fonds

du Gouvernement ? Nous considérons que cet amendement est satisfait, puisque le projet régional de santé intègre obligatoirement les objectifs portant sur la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Comme vient de le rappeler M. le rapporteur

Dans la suite de notre débat sur la nécessité de mieux représenter les élus dans les conseils d'administration des ARS, nous proposons de renforcer les pouvoirs de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, d'abord, faire en sorte qu'elle donne un avis conforme, et pas seulement consultatif, sur le projet régional de santé ; ensuite, qu'elle soit informée régulièrement, par le directeur général de l'ARS, de la mise en oeuvre du projet régional de santé et des moyens qui sont concrètement attribués aux territoires ; enfin, qu'elle dispose d'un budget propre pour mener sa propre expertise et ses propres initiatives. Chacun le sait, il existe de nombreux collèges dans la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, ainsi qu'une forte représentation des élus locaux de l'ensemble des collectivités. Il nous semble que ce lieu de coélaboration pourrait être rénové.

de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin n'est pas une agence régionale, c'est pour prendre en compte les statuts des trois collectivités de son ressort. La Guadeloupe est, en effet, un département-région régi par l'article 73 de la Constitution, quand Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution. La rénovation de la gouvernance des agences régionales transformant le conseil de surveillance en conseil d'administration doit donc traduire cette diversité statutaire. Le président de la région Guadeloupe ne peut pas participer à cette instance au nom de la collectivité de Saint-Barthélemy, ni de la collectivité de Saint-Martin. Par ailleurs, Saint-Barthélemy est en dehors du ressort de la région de Guadeloupe et exerce pleinement les compétences régionales. Elle est donc légitime à siéger au conseil d'administration de l'Agence de santé, au même titre que n'importe quelle région. À la faveur de cette évolution, l'article 31 attribue, en outre, au conseil d'administration des compétences telles que l'approbation de la politique de contractualisation avec les collectivités. Ce qui pouvait se concevoir pour un conseil de surveillance se conçoit moins pour un conseil d'administration. Le premier se bornait à approuver les comptes de l'agence et à émettre un avis simple à la majorité simple, sur le projet régional de santé. De plus, la crise sanitaire a mis en lumière la nécessité de territorialiser davantage la politique sanitaire, supposant une plus grande implication des élus. La collectivité de Saint-Barthélemy est un acteur de la politique sanitaire. Elle a ainsi très tôt pris l'initiative et financé la définition d'un protocole sanitaire, acquis du matériel pour la réalisation de tests et des respirateurs. Elle met notamment gracieusement à disposition de l'hôpital la cuisine et la buanderie de l'Ehpad. Elle loge une partie du personnel de l'hôpital et apporte sa garantie financière au groupement de coopération sanitaire abritant un scanner, un mammographe et une table de coronarographie. Cela permet d'alléger le coût de la politique sanitaire, car chaque examen effectué à Saint-Barthélemy permet à la sécurité sociale de ne pas avoir à supporter le remboursement du trajet vers Saint-Martin. Pour ces raisons, la gouvernance du conseil d'administration doit refléter la réalité territoriale de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'amendement : La parole est à M. le rapporteur. Le texte issu des travaux des commissions a prévu la coprésidence du conseil d'administration des ARS par le président du conseil régional ou son représentant, aux côtés du préfet de région. Une coordination est toutefois nécessaire à l'article L. à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique relatif à l'agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, qui exerce, dans ces territoires, les compétences dévolues aux ARS. Le conseil de surveillance de cette agence de santé est présidé, aux termes de cet article, par le représentant de l'État en Guadeloupe. Il est donc proposé que cette instance, transformée en conseil d'administration par le projet de loi, soit coprésidée par le président du conseil régional de Guadeloupe ou son représentant.

de proposer une coordination pour la coprésidence du conseil administration de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Celle-ci est actuellement présidée par le représentant de l'État en Guadeloupe ; il me semble donc plus cohérent d'en confier la coprésidence au président de la région Guadeloupe.

toute leur place dans la composition de ce conseil, au titre des représentants des collectivités territoriales. Le principe de vice-présidence, qui pourra être prévu, comme à l'heure actuelle, au niveau réglementaire constitue probablement une réponse plus pertinente.

car on s'aperçoit que, malgré tout, l'essentiel des décisions remonte au niveau ministériel, ce qui ne constitue pas un bon principe de fonctionnement. On a voulu ces agences régionales de santé, il est donc important qu'elles puissent fonctionner en toute autonomie, d'autant plus que

De la même manière que le directeur général de l'ARS est tenu de rendre compte à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, il serait ainsi tenu de présenter le bilan de ses actions aux conseils départementaux, afin de fluidifier les relations entre les ARS et les conseils départementaux. Certains directeurs d'ARS nous ont sollicités et ont manifesté leur volonté de renforcer les liens et les échanges entre l'ARS et les conseils départementaux.

Lors de plusieurs auditions, il a été porté à notre attention un manque de relation entre les représentants de l'ARS et les élus locaux, malgré les mesures actuellement en vigueur. Nombreux sont ceux qui nous ont fait part d'un problème d'information, d'une part, et du peu d'échanges avec l'ARS,

était soit faible, soit très faible. Il apparaît donc que le simple partage de bilan ne suffit pas. L'envoi de ces documents ne répond pas efficacement au besoin d'information. C'est pourquoi il nous apparaît pertinent de proposer de l'ARS, ou son représentant, soit invité à rendre compte de la politique de santé sur le territoire, afin non seulement de permettre un temps d'échange, mais également d'assurer un suivi et de créer une relation entre les élus locaux et l'ARS. Quel est l'avis de la commission

est à M. Thomas Dossus. La pandémie en cours met en lumière de façon éclatante le besoin d'adhésion et de participation de la population aux politiques de santé publique. Les politiques publiques verticales

les conseils territoriaux de santé et les contrats locaux de santé. Les conseils territoriaux de santé regroupent les acteurs de la santé d'un territoire. Leur rôle est de réaliser des diagnostics afin de définir une meilleure politique locale sur un territoire. Ils organisent déjà l'expression des usagers, mais dans une formation spécifique. Nous souhaitons renforcer ce lien avec les usagers, en affirmant que les CTS « garantissent la participation » des usagers

s'agissant des contrats locaux de santé. Ces contrats, conclus entre les ARS et les collectivités, visent à réduire les inégalités éventuelles de la politique régionale de santé en prenant en compte la spécificité des territoires, notamment les zones périurbaines et rurales. que ces contrats garantissent la participation des usagers- de tous les usagers. Comme dans tous les domaines, une décentralisation en matière de santé ne peut être réussie que si elle associe étroitement les premiers concernés. Quel

Mme Raymonde Poncet Monge. En matière de santé, c'est la prévention qui prime. Une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation, un accompagnement social et médical efficace et de proximité permettent de réduire les maladies. La France s'est dotée de dispositifs de prévention en santé relativement efficaces. Par exemple, le volet « prévention » de la stratégie nationale de santé présentée en 2018 par Mme Buzyn comportait un large éventail d'actions de prévention bienvenues.

En cohérence avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales ont une responsabilité essentielle pour mettre en oeuvre des politiques efficaces de prévention en matière de santé environnementale.

dont la mienne, l'Auvergne-Rhône-Alpes ; cinq autres obtiennent à peine la moyenne, et seule une région est saluée pour la qualité des mesures engagées. Il faut rehausser nos objectifs. L'environnement est l'un des premiers responsables de la survenue de maladies chroniques.

particulièrement efficace dans la lutte contre l'épidémie. Cet amendement a donc pour objet de généraliser la conclusion de contrats locaux de santé sur l'ensemble du territoire national. Nous l'avons déjà dit, les territoires jouent un rôle indispensable dans les politiques de santé publique, notamment par leur coordination des acteurs de la ville et hospitaliers. En réalisant un diagnostic des objectifs partagés, les contrats locaux de santé sont une réponse au besoin d'articulation et de cohérence entre l'action nationale et locale. À ce titre, ils doivent être encouragés et généralisés. C'est pourquoi le présent amendement, porté par Jean-Pierre Corbisez, vise à généraliser ce dispositif sur l'ensemble du territoire, afin que chaque territoire bénéficie d'un cadre de dialogue et d'action partagés avec l'État.

régionales de santé et nos collectivités est porteur de politiques de santé territorialisées et adaptées, lesquelles sont précieuses, notamment, pour les zones rurales isolées et les quartiers urbains en difficulté. Il est toutefois regrettable que les maladies mentales et les troubles psychiques n'y soient pas systématiquement identifiés comme l'un des axes majeurs de notre politique sanitaire. La crise du covid 19 que nous traversons a tristement mis en lumière la détresse de certains de nos concitoyens ; je pense notamment à nos jeunes étudiants, particulièrement éprouvés. des initiatives locales isolées ont pu voir le jour, la santé mentale nécessite une action coordonnée de l'État et des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités. C'est pourquoi cet amendement

suicides des étudiants et les alertes des pédopsychiatres nous imposent de prendre la mesure de l'urgence. La santé mentale est malheureusement le parent pauvre des politiques de santé publique. Seuls 40 % des personnes souffrant de troubles psychiques sont aujourd'hui prises en charge, pour des questions complexes d'acceptation sociale de ces maladies, certes, mais aussi et surtout à cause de réelles difficultés d'accès aux soins. Nous devons nous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Ainsi, en 2010, l'Australie a lancé le programme santé mentale,

Comme vient de le rappeler ma collègue, le suicide est la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans. La pandémie a encore aggravé la situation. En faisons-nous assez face à ce fléau sociétal ? Peut-on s'exonérer de cette problématique ? Ce sujet criant doit nous interpeller. La santé mentale nécessite une action coordonnée de l'État et des autorités sanitaires, des associations de soutien et de prévention et des collectivités.

Je suis d'accord avec les auteurs de ces amendements : la santé mentale est un enjeu majeur, qui mérite d'être pris en compte dans les politiques territoriales de santé. Toutefois, c'est déjà le cas. Je rappelle que nous avons mis en place les projets territoriaux de santé mentale, qui sont en cours d'élaboration.

permettre de jouer un rôle d'ensembliers et de facilitateurs et d'organiser la convergence avec les politiques publiques mises en oeuvre sur le territoire et concourant au renforcement de la santé globale de la population. Le présent amendement tend donc à prévoir que toute collectivité ou tout groupement signataire d'un contrat local de santé dispose d'un siège au sein du conseil d'administration de la CPTS, située en tout ou partie sur le territoire du CLS.

Porteurs d'actions concrètes et directes au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations, ils sont en mesure d'intervenir sur l'ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé. À ce titre, les communautés professionnelles territoriales de santé sont des acteurs essentiels de la santé sur le territoire. Afin de soutenir au mieux les acteurs de santé, de faciliter leur coordination et de renforcer le maillage sanitaire sur le territoire, une discussion est nécessaire sur le périmètre de déploiement des CPTS, en des CPTS, en cohérence avec l'existence de contrats locaux de santé ou de tout autre dispositif territorialisé d'accès aux soins et de prévention. Le présent amendement tend ainsi à proposer que, lors de l'élaboration d'une CPTS, son périmètre puisse être transmis aux collectivités et aux groupements signataires de contrats locaux de santé, afin qu'ils puissent exprimer un avis sur la meilleure manière d'articuler ces initiatives.

Ils sont porteurs d'actions concrètes et directes, dans le champ de leurs compétences et par leurs actions, au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leurs populations. Ils sont en mesure d'intervenir sur l'ensemble des déterminants sociaux et environnementaux de santé- qualité de l'eau, qualité de l'air, expositions, nuisances sonores, habitat. Par ailleurs, ils jouent un rôle déterminant d'ensembliers pour coordonner les acteurs de la ville et de l'hôpital sur leurs territoires, comme l'a montré la crise sanitaire. sanitaire. Le présent amendement tend à prévoir que lors de l'élaboration d'une CPTS, son périmètre puisse être transmis aux collectivités et aux groupements signataires de contrats locaux de santé, afin qu'ils puissent donner leur avis sur la meilleure manière d'articuler ces initiatives indispensables avec les espaces de dialogue déjà existants.

dans la mesure où ces communautés ont d'abord vocation à permettre aux professionnels de santé une meilleure coordination de leur action pour concourir à la structuration du parcours de soins et du parcours de santé. Cet outil doit rester à la main

est la plus forte en France. Le dernier recensement a eu lieu en 2017, mais une augmentation encore plus importante est à prévoir dans ce territoire, où le taux de natalité est trois fois supérieur à celui de l'Hexagone. Enfin, la topographie de l'île rend l'accès à ces officines difficiles pour nombre d'habitants. Il apparaît donc que les critères actuels ne permettent pas de répondre efficacement aux spécificités du territoire de Mayotte.

De plus, les conditions démographiques exigées pour l'ouverture d'une officine doivent être remplies depuis deux ans à compter de la publication du dernier recensement. La conjonction de ces deux critères est un véritable frein au développement du réseau officinal dans le département de Mayotte.

le délai de deux ans à compter du recensement général attestant que les seuils démographiques sont atteints

Nous voulons ainsi garantir une représentation complète et plurielle, mais également assurer une meilleure représentation des élus territoriaux dans leur diversité politique et leur diversité locale, en prévoyant notamment la présence d'élus de territoires ruraux. Quel

En revanche, nous n'avons pas considéré comme opportun d'introduire par la loi la présence d'élus nationaux dans une instance au sein de laquelle sont déjà représentés des élus locaux, conformément à la volonté de

en leur permettant d'intervenir dans l'organisation du travail. Nous souhaitons créer un comité territorial des élus participant à l'élaboration des projets régionaux de santé. Il nous semble indispensable de prévoir, à tous les échelons décisionnels, une augmentation du nombre de représentants dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets territoriaux de santé. Dans un souci de proximité, l'élaboration du diagnostic territorial partagé, qui sert de fondement à l'élaboration des projets territoriaux de santé, nécessite de prévoir une concertation avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L'amendement

Alors que les membres du troisième collège sont actuellement désignés, pour trois d'entre eux, par le représentant de l'État, et, pour deux d'entre eux, par le directeur de l'agence régionale de santé, l'ARS, il est proposé qu'un des cinq membres soit désigné par le représentant de l'association des maires du département d'implantation de l'établissement hospitalier. Enfin, le président du conseil de surveillance serait désigné uniquement parmi le collège des élus.

opportun de revenir sur l'équilibre entre les trois collèges, élus locaux, personnels de l'hôpital et personnalités qualifiées, composant ce conseil de surveillance. Les collectivités demeurant un financeur subsidiaire des établissements publics de santé, je ne trouve pas pertinent de revenir sur l'équilibre actuel, qui permet déjà de leur assurer une place dans ces instances. Par ailleurs, la rédaction actuelle du code de santé publique n'exclut pas la participation au conseil de surveillance d'élus régionaux.

la question de l'implantation des médecins en particulier. Établi conjointement avec le groupe d'études développement économique de la montagne, et sur la base de la proposition de loi n° 681 visant à lutter contre les déserts médicaux, cet amendement a pour objet de mettre en place des commissions départementales de démographie médicale composées de représentants de l'État, de l'ARS, des collectivités territoriales et des membres du conseil départemental de l'ordre des médecins. Ces commissions seraient chargées de définir les projets territoriaux de santé, les contrats territoriaux de santé et les projets d'aire de santé et d'approuver les projets de création de pôle de santé et de maisons de santé, afin de répondre au mieux aux besoins des territoires et de la population.

les stages des étudiants en fin d'année de médecine, le principe de convention sur ce sujet entre l'assurance maladie et les représentants des médecins. Toutefois, le principe des commissions départementales que l'amendement vise à instituer appelle plusieurs réserves. d'abord, la notion d'« aire de santé » se superposera aux zonages établis par les ARS en liaison avec les professionnels de santé, ce qui ne participe pas de la bonne visibilité d'ensemble de ces dispositifs déjà complexes à appréhender par les acteurs de terrain. Ensuite, vous n'évoquez que la démographie médicale alors que les coopérations entre professionnels de santé sont une piste intéressante pour améliorer l'accès aux soins dans les territoires. Enfin, il existe déjà de nombreuses données de diagnostic sur l'état de la démographie médicale. Plusieurs structures existent au niveau territorial, dont les conseils territoriaux de santé, que vous évoquez. Je ne pense pas que la création d'une nouvelle structure, départementale, et d'un nouveau dispositif, les aires de santé, apportera une réponse opérationnelle aux besoins de nos concitoyens. Il me semble plus efficace de poursuivre les efforts engagés pour créer des conditions de travail attractives pour les professionnels de santé : exercices en en équipe et coordonnés, notamment les maisons de santé ; possibilité d'exercice mixte ville-hôpital ; simplification et appui, par exemple le déploiement d'assistants médicaux pour permettre aux médecins de se recentrer sur leur coeur de métier. Par conséquent, à défaut d'un retrait

selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la Drees. En outre, les budgets de l'hôpital public sont en baisse de 10 % sur dix ans.

permettant aux collectivités de financer elles-mêmes les établissements de santé que l'on parviendra à un rééquilibrage ; cela risque au contraire d'accroître les inégalités.

sur les finances des collectivités territoriales. C'est d'ailleurs l'une des réserves que j'ai exposées sur cet article, qui ne doit pas conduire à une aggravation des inégalités territoriales en matière de santé. C'est pour cela que j'ai proposé une modification de la rédaction de l'article visant à insister sur la notion de « concours Plusieurs lacunes sont aussi à signaler. Il me semble préjudiciable de remplacer le programme d'investissement défini dans le code de santé publique par la notion de « projet ». Surtout, il est proposé de mentionner les communes dans chacun des articles codifiés, dont ceux qui concernent les départements et les régions.

Cet amendement, déposé sur l'initiative de notre collègue Philippe Mouiller, vise à associer les représentants des collectivités territoriales à la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, ainsi que les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé. répond à l'objectif qui figure dans l'étude d'impact du projet de loi : adapter l'offre de soins aux besoins identifiés sur chaque territoire. À l'heure actuelle, le directeur général de l'ARS détermine les zones blanches médicales après concertation avec les représentants de chaque profession de santé concernés, et après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Cette conférence comporte, certes, un collège d'élus, mais ceux-ci ne représentent que dix membres parmi une centaine. Ce zonage, dans la détermination duquel les élus ne sont donc impliqués que de manière très résiduelle, conditionne toutefois l'aide susceptible d'être apportée par une collectivité territoriale à une structure de soins.

L'article L. 1434-4 du code de la santé publique prévoit une définition de ces zones en concertation avec les professionnels de santé concernés.

Nous pensons que cet article est un aboutissement, puisqu'il permet d'inscrire dans le droit une évolution malheureusement devenue nécessaire : la création de centres de santé gérés par la puissance publique.

Aujourd'hui, il va même investir pour améliorer les locaux. J'ai travaillé avec M. le préfet du Pas-de-Calais sur la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, dans le département pour inclure la notion de soutien aux centres de santé, et non plus aux seules maisons de santé. Cela reste un souci.

les pôles métropolitains, les agences départementales, etc. Par conséquent, nous proposons de la remplacer par les termes « les établissements publics de coopération intercommunale ».

n° 660 rectifié. En limitant la possibilité de créer des centres de santé aux seuls départements, communes et EPCI, l'article 34 a pour effet de priver les régions de cette faculté. certaines d'entre elles se sont particulièrement investies pour favoriser l'accès aux soins de leur population, en se fixant par exemple comme objectif de créer des postes de médecins salariés. De surcroît, en excluant les régions de ce dispositif, les politiques de soutien qu'elles conduisent en faveur de la mise en place de tels centres s'en trouveront fragilisées du fait de la suppression de leur clause de compétence générale. Aussi, le présent amendement de mon collègue Jean-Pierre Corbisez vise à rétablir cette possibilité pour les régions.

a pour objet d'harmoniser les dispositions des articles 33 et 34 du projet de loi. L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique dispose que les EPCI peuvent créer et gérer des centres de santé, alors que l'article 34 adopté par la commission des lois ouvre cette faculté aux groupements de collectivités. La notion de groupements de collectivités est une acception qui nous semble trop large. Par conséquent, il est proposé de maintenir cette faculté pour les seuls EPCI.

présenter l'amendement n° 798 rectifié. La politique de santé relève de la responsabilité de l'État. Sans remettre en cause le caractère régalien de cette compétence, il importe de tirer les enseignements de la crise, en reconnaissant dans leurs champs de compétences et dans leurs actions, les territoires contribuent directement à la conception d'un écosystème global de santé. Ils doivent donc être considérés comme des interlocuteurs privilégiés de l'État, lorsque celui-ci élabore et conduit sa politique sanitaire. Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler cet état de fait, particulièrement visible durant la crise sanitaire. Logement, mobilité, les collectivités sont des productrices de santé globale et doivent donc être consultées et associées par l'État, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé et, comme nous l'avons vu durant la crise épidémique, de préparation et de réponse aux crises sanitaires.

doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne et que les professionnels, les établissements de santé, les organismes d'assurance maladie et les autorités sanitaires contribuent à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Garantir l'égal accès aux soins, n'est-ce pas justement une disposition politique que portent particulièrement les collectivités territoriales ? Les territoires sont des acteurs incontournables des politiques publiques de santé, en particulier dans le champ de la prévention. Ils sont porteurs d'actions concrètes, directes, au bénéfice du bien-être physique, social et mental de leur population, au travers des politiques d'accès au soin et d'accompagnement social. De même, la crise sanitaire a démontré l'importance fondamentale de l'implication des départements, des régions et des communes dans la gestion des réponses sanitaires d'urgence. Ce sont les collectivités qui, massivement, ont fourni des équipements de protection individuelle et des masques, lorsque le stock stratégique de l'État, non

proximité qui mobilisent leurs moyens financiers, logistiques et humains. Dès lors, pourquoi ne sont-ils pas cités parmi les organismes qui contribuent à la mise en oeuvre de la protection de la santé ? Cet amendement vise à pallier cet oubli,

Genet, pour présenter l'amendement n° 797 rectifié. Sans demander de nouvelles responsabilités sanitaires pour les collectivités et leurs groupements, cet amendement vise à rappeler le rôle des territoires, particulièrement visible durant la crise sanitaire. Logement, mobilité, eau, air ... les collectivités sont des productrices de santé globale et doivent donc être consultées et associées par l'État, notamment en matière de promotion de la santé, de parcours de santé et, comme nous l'avons vu durant la crise épidémique, de préparation et de réponse aux crises sanitaires. Cet amendement vise donc à reconnaître le rôle assumé par les territoires, ainsi que la nécessité d'un dialogue étroit avec l'État.

cet amendement permettrait à la Ville de Paris d'expérimenter une organisation administrative plus souple au sein de ces services, pour bien distinguer les missions de PMI qui relèvent de la petite enfance et celles qui relèvent de faire en sorte que la hiérarchie exercée par le médecin-chef de la Ville ne concerne plus que les activités de santé et ne soit plus obligatoire pour les activités de petite enfance.

de la santé avec celles qui sont relatives à l'accueil de la petite enfance. Il s'agit dès lors de structurer une équipe dédiée à l'agrément des modes d'accueil, des assistantes maternelles et des assistants familiaux et de concentrer l'action des professionnels de santé du service de PMI sur leurs missions plus directement liées à la santé.

dans l'exercice de ses missions, que les missions d'agrément s'exerceront sous l'autorité fonctionnelle du médecin-chef de service de la protection maternelle infantile qui pourra déléguer les missions correspondantes au responsable du service en charge de l'agrément des modes d'accueil. Quel

qui concerne l'expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active,

avec quelques départements volontaires, le transfert à l'État de l'instruction administrative, de la décision d'attribution et du financement du RSA et du revenu de solidarité, de manière à mettre un terme aux difficultés chroniques

Le groupe écologiste n'est pas opposé à l'expérimentation de la recentralisation sur une base volontaire, mais force est de constater que la motivation principale, sinon unique, unique, est bien financière, la part de cette dépense dynamique supportée par les départements devenant, pour certains, ingérable dans le cadre d'un budget contraint. en est une participation insuffisante de l'État à cette prestation universelle, qui, dès lors, conduit à comprimer les budgets dédiés à l'accompagnement des allocataires, alors même que son montant est nettement insuffisant et exclut les jeunes de moins de 25 ans. Le reste à charge pour les départements est de 4 milliards d'euros, mais la progression inédite en 2020, du fait de la crise sanitaire et sociale, touche les départements de façon différenciée. Certains attendent de la recentralisation, tout simplement, un allégement du poids financier, l'État prenant enfin, par cette voie,

La recentralisation doit permettre aux départements de consacrer plus de moyens à l'accompagnement social et à l'insertion, qui restent ses véritables compétences. Dès lors, il conviendra de veiller aux ressources fléchées vers cette action sociale. ailleurs, cette recentralisation ne saurait accompagner un renforcement de la politique de contrôle, voire de double contrôle : ce serait un comble alors que l'on mesure déjà les effets délétères d'une perte de bienveillance envers ce public des plus précaires, à qui il faudrait avant tout redonner confiance. C'est la conséquence d'un discours, martelé sans cesse, appelant à toujours plus de contrôle social. Plus de capacité d'accompagnement et de soutien par des travailleurs sociaux de proximité